L'objet de l'article 15 est d'étendre ces dispositifs de réassurance de la caisse centrale de réassurance aux grandes entreprises et aux risques d'assurance-crédit à l'export. Aujourd'hui, seules les entités françaises d'une entreprise française Je vous remercie

La délégation de service public à des filiales peut s'avérer pertinente dès lors qu'elle permet davantage de souplesse et de proximité dans la mise en oeuvre des actions publiques. Nous partageons bien sûr ce point de vue et la logique de cet article, mais le risque existe que cette délégation de service public complexifie le contrôle réalisé par le Parlement sur l'emploi des ressources publiques. par cet amendement, que les filiales rendent compte au Parlement des actions qu'elles mènent au nom de l'AFD. Cela permettra notamment aux membres des commissions des finances d'interroger le directeur de l'AFD sur l'utilisation de cet argent public sur la base d'éléments concrets. Il s'agit là de renforcer le rôle du Parlement.

Garriaud-Maylam. Il y a longtemps que les Français de l'étranger s'interrogent sur le soutien aux petites entreprises françaises. Lors d'une réunion de la commission des affaires étrangères, j'avais interrogé le président de l'AFD à ce sujet et lui avais demandé qu'un soutien soit apporté par son agence aux

probablement dans l'idée d'aider les PME françaises installées et enregistrées en Afrique, ce dispositif est encore

de vote. Je partage ce qui vient d'être dit par mon collègue Leconte : bien évidemment, cet avis défavorable est absolument incompréhensible. Cela va totalement à l'encontre des intérêts français à l'étranger et de ceux de nos petites entreprises, qui contribuent à notre commerce extérieur

et, surtout, nos collègues- puisque ce sont eux qui voteront en leur âme et conscience -que nous devons vraiment poser un acte de solidarité envers ces petits entrepreneurs qui, encore une fois, contribuent au rayonnement de la France et à notre commerce extérieur. La parole

etc., des actifs immobiliers qui contribuent à l'économie réelle- des commerces, des usines, des appartements servant à héberger

Il demeure le dernier dispositif- et sûrement le plus opérationnel et le plus simple -pour accompagner l'investissement forestier. Il est donc important de le reconduire, tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace.

3 sont fondés sur la dette, je pense notamment aux prêts garantis par l'État, les PGE : 300 milliards de crédits possibles ont été ouverts. C'est très bien, cela permet de soutenir les entreprises pendant la crise, mais il existe un énorme problème de fonds propres.

a trois conséquences pour le marché de la musique enregistrée : une baisse de 20 % des ventes par rapport au prévisionnel pour 2020, une hausse des charges liées aux multiples reports et annulations et, enfin, un impact en partie différé du fait de l'effondrement des droits voisins qui se traduira par une baisse de revenus et une attrition des aides à la création servies par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir. La crise sanitaire vient donc ébranler un marché fragilisé par quinze ans de crise des supports physiques. Or dans une économie de prototype, comme celle de la musique enregistrée, la reprise dépendra de la capacité des entreprises à continuer à prendre des risques dans un environnement malheureusement dégradé. Cet amendement tend donc à prévoir une hausse temporaire des taux pour les années 2020 à 2024 afin d'accompagner la reprise. Il tend également à faire passer le taux TPE-PME de 30 % à 40 % et les taux des autres entreprises de 15 % à 25 %, ce qui permet de maintenir des taux différenciés selon la taille des entreprises tout en soutenant l'ensemble du secteur, la crise affectant des répertoires musicaux défendus indifféremment par des petites ou des moyennes entreprises. Renforcer le CIPP maintenant, c'est permettre aux labels de continuer à investir dans la production de nouveaux talents francophones- j'insiste qui est la partie de leur activité à la fois la plus risquée, mais aussi la plus essentielle au regard de la diversité des esthétiques.

vise à porter de 1,1 à 2 millions d'euros le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l'État : 1 euro de crédit d'impôt investi représente en moyenne

autres États membres. Il s'agit, d'une part, de soutenir le réseau de distribution de la musique qui a subi un recul de près de 10 % par an sur les cinq années avec la montée en puissance du et, d'autre part, de soutenir l'activité des labels très dépendants du marché physique alors que le confinement a été brutal et immédiat pour ce segment.

Cette certification est l'un des leviers importants pour promouvoir l'agroécologie et la montée en gamme de notre agriculture. Elle a été créée il y a maintenant dix ans, à l'occasion du Grenelle de l'environnement.

Mme la ministre déléguée. Il s'agit de supprimer l'article 16 du présent projet de loi de finances rectificative, qui inclut le théâtre dans le champ du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants. En l'état, les paramètres du dispositif ne sont pas adaptés aux spécificités propres au secteur du théâtre. Le crédit d'impôt « spectacles vivants » a pour objectif de soutenir la production d'artistes émergents dans le domaine musical et d'accompagner des entreprises moins subventionnées et prenant des risques financiers. Il a été conçu pour accompagner des artistes qui ont dû faire face à la crise du disque et qui ont dû se reporter sur les tournées, comme vous l'avez mentionné à propos du crédit d'impôt phonographique. Conscient des difficultés que rencontre le secteur du théâtre dans le contexte de la crise sanitaire, le Gouvernement s'engage à retravailler une proposition et à proposer une mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Vous savez d'ailleurs que la ministre de la culture a été très claire sur ce sujet.

ces deux composantes du spectacle vivant de côté. Si nous voulons voir l'économie de la culture, tout particulièrement celle du spectacle vivant, redémarrer en ces temps difficiles, nous devons faciliter l'investissement pour les entrepreneurs de la filière.

tout récemment, au-delà des différences politiques, pour inscrire les articles 16 et 16 dans ce PLFR. Aujourd'hui, les entreprises du spectacle et les artistes nous observent. Il faut rejeter ces amendements de suppression du Gouvernement pour que les deux articles mentionnés soient votés conformes dans les deux chambres. Je mets aux voix

a évalué pour le secteur la baisse moyenne du chiffre d'affaires à au moins 25 % en 2020, soit un recul à attendre de plus de 22,3 milliards d'euros. Le poids économique de la culture, c'est près de 79 800 entreprises et 635 700 emplois directs. Le spectacle vivant est en première ligne des difficultés, après le cinéma et l'audiovisuel. Les annulations de festivals et de rencontres estivales partout en France mettent en sommeil le secteur pour de longs mois. Afin de le relancer et de contribuer au maintien de la diversité culturelle française, sur notre territoire et au-delà, l'amendement vise à dynamiser le CISV avec une bonification des taux en 2020 et en 2021, avant un retour progressif au taux de 2019 les années suivantes. Il est également proposé d'augmenter les plafonds par projet et par entreprise pour aider les entreprises à supporter les coûts engagés pour les événements annulés ou reportés, et leur permettre également de développer de nouveaux projets. La parole

ou à un autre. Dix ans après l'application au livre audio d'un taux réduit de TVA de 5,5 %, le présent amendement vise à appliquer ce même taux aux produits physiques musicaux relevant d'un acte d'achat- ventes de CD, vinyles et téléchargements -à compter du 1 janvier 2022,

En 2020, on estime à 156 millions d'euros les pertes de chiffre d'affaires pour ce seul segment par rapport au prévisionnel pré-crise. Cette mesure historique bénéficierait également à l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris au public qui manifeste chaque année son attachement aux artistes de la scène française : 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français. Dans un marché avec une telle dominante tricolore, le risque d'effet d'aubaine au profit des productions étrangères est totalement écarté.

Cadic. Lorsqu'une entreprise fait un don à un organisme d'intérêt général, elle bénéficie d'une réduction d'impôt imputable sur les bénéfices réalisés par l'entreprise pendant cinq ans.

Financement la mise en oeuvre de deux dispositifs de prêts aux entreprises créés par la dernière loi de finances rectificative : l'octroi à de petites entreprises de prêts participatifs financés sur le fonds de développement économique et social, et l'octroi d'avances remboursables et de prêts bonifiés aux PME. Cet article vise, d'autre part- et c'est important par rapport à la question des besoins en fonds propres -, à étendre le bénéfice de ce dispositif d'avances aux entreprises de taille intermédiaire. Je précise que les avances remboursables sont regardées comme des quasi-fonds propres. Quel est l'avis de

: La parole est à M. Vincent Segouin. Cet amendement vise à ce que les prêts garantis par l'État puissent être classés dans les fonds propres des entreprises, à hauteur de la garantie de l'État, plutôt que dans les dettes.

l'Assemblée nationale, vise à obliger les banques à notifier par écrit leur refus d'octroyer un prêt garanti par l'État aux entreprises. En l'état actuel de la rédaction, ce délai consenti aux banques doit être « raisonnable Cette rédaction imprécise laisse une large place à l'interprétation. Or on peut légitimement s'attendre à ce que les banques refusant le prêt, d'une part, et les entreprises l'ayant demandé, d'autre part, n'en aient pas la même interprétation. Aussi, afin de limiter le nombre de contentieux, de préciser le texte de la loi, de sécuriser le dispositif et de mieux répondre à l'objectif affiché, à savoir permettre aux entrepreneurs de se tourner rapidement vers d'autres solutions de financement, cet amendement vise à fixer ce délai à cinq jours, un délai à la fois raisonnable et précis.

Nathalie Goulet. Cet amendement est proposé par Sylvie Vermeillet. L'arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, élargit la possibilité de recours au dispositif de prêt garanti par l'État (PGE) pour les entreprises en difficulté qui font l'objet d'une procédure collective depuis le 1 janvier 2020. Le présent amendement vise à élargir le bénéfice du PGE aux entreprises qui faisaient déjà l'objet d'une procédure collective avant le 1 janvier 2020 et la survenance de la crise liée au coronavirus.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement, proposé par Claude Kern, tend à mettre en place un dispositif exceptionnel, sous condition de revenus, de crédit d'impôt pour la délivrance et le renouvellement de licences sportives dès publication de la loi et jusqu'au 31 décembre 2020. Cela permettra aux associations sportives, durement touchées par la crise sanitaire, de reprendre pleinement leurs activités à la rentrée de septembre, en permettant également aux familles de gérer leurs autres priorités. Quel

incitées à mettre en place cette exonération, ainsi que de la concurrence entre des collectivités locales dont les situations peuvent être très différentes. Plutôt que de baisser encore les ressources des collectivités locales sans relancer le tourisme, autant supprimer ce mécanisme d'exonération facultatif.

décidées par délibération des collectivités locales ne me posent pas de difficultés sur le plan des principes, et je suis pour la liberté. Après tout, si une commune veut mettre en place telle ou telle exonération,

L'article 17 vise à permettre aux communes et EPCI de décider des exonérations de taxe de séjour en 2020 pour les entreprises de leur territoire. Cette mesure serait salutaire pour préserver, à la fois, le tissu des entreprises locales et l'attractivité des territoires. En l'état actuel, cette décision doit intervenir avant le 31 juillet 2020. Compte tenu du calendrier des élections propres au bloc communal, d'une part, et du calendrier législatif, d'autre part, ce délai paraît beaucoup trop contraint pour espérer que les communes et les EPCI se saisissent, entre la date de promulgation de la loi et la fin du mois de juillet, de ce levier d'action en faveur de l'économie des territoires. J'invite mes collègues qui ont adopté un amendement similaire visant au dégrèvement de la à voter de façon cohérente, afin que le bloc communal puisse prendre de telles décisions dans des délais raisonnables, en repoussant cette date du 31 juillet au 30 septembre. Quel est l'avis de la

de gérer. On a repoussé de nombreuses dates, mais, à un moment, il y a une limite à ce que peuvent faire les services de la direction générale des finances publiques afin de sécuriser ces exonérations.

indirects et obligatoires, sur les causes qui leur sont chères. Cela permettrait de maintenir la collecte en faveur des associations, notamment dans le domaine social, et d'indiquer aux donateurs non imposables que leur don, quel qu'en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables.

J'émets également un avis défavorable.

permanente, totale ou partielle, au profit des entreprises exerçant une activité en zone extracommunautaire et qui implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. Il s'agit donc

qui le souhaitent de participer à l'effort de rapatriement des chaînes de production sur le territoire, pour remédier aux ruptures d'approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale.

Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies sur les récoltes forestières. les coupes de bois ne s'opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers et il est souvent difficile d'apprécier l'impact d'un sinistre dans les quinze jours où il survient. L'épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité associée au scolyte typographe, en est un parfait exemple. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit, à ce jour, le 31 décembre de l'année suivante.

Cette exonération existe déjà pour les disquaires indépendants, qui facilitent l'accès à la culture sur notre territoire. Une extension aux petits éditeurs de musique dans le contexte de la reprise contribuerait à soutenir la création musicale. Dans cette perspective, la mesure d'exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à abaisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur.

Il s'agit de revenir sur la réforme de la retenue à la source pour les personnes non résidentes. En effet, cette réforme conduirait un certain nombre de non-résidents

parce que, en exonérant du forfait social la part de la participation excédant la formule légale pour les PME et les ETI, vous n'incitez pas ces entreprises à conclure de tels accords, puisqu'elles sont déjà dans l'obligation de prévoir un dispositif de participation. Finalement, cela créerait un effet d'aubaine, puisque la participation est obligatoire et que l'on ne parle pas d'intéressement. Or ce qui nous intéresse, c'est de développer d'autres formules de partage de la valeur et d'association des salariés à la réussite de l'entreprise.

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à prolonger le dispositif adopté dans la deuxième loi de finances rectificative pour inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus par les entreprises locataires

Le présent amendement vise à inclure dans le champ du crédit d'impôt les filiales des éditeurs de services de télévision dont l'objet social exclusif est de procéder à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques.

L'article 17 crée un nouveau crédit d'impôt pour soutenir la création audiovisuelle et cinématographique. Il s'agit d'un effort réalisé par la collectivité pour soutenir la création artistique en France. Pour rappel, aucune étude d'impact n'a été réalisée, puisque cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il convient de restreindre le dispositif à sa vocation de soutien aux activités culturelles sur le territoire national et de trouver un équilibre entre responsabilité budgétaire et incitation fiscale. C'est l'objet de cet amendement, qui tend à exclure du crédit d'impôt les dépenses qui seraient réalisées hors de France, afin de concentrer les efforts sur les dépenses qui bénéficieront à l'économie nationale.

La séance est reprise.

dont bénéficient les associations foncières pastorales. Cette exonération a été mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises. Au regard des retombées très positives qu'apportent ces associations sur les plans environnemental et économique, il est proposé de la reconduire pour trois années supplémentaires. Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Ainsi, le coût total de cette mesure s'élève à environ 50 000 euros sur l'ensemble du département de l'Ariège. Cependant, ce dispositif représente une contrepartie réelle et appréciée, qui permet de faciliter l'action publique de dynamisation des territoires ruraux de montagne. L'activité pastorale dans nos montagnes favorise l'activité économique et sociale, et le maintien des services publics dans nos vallées. L'adoption de cet amendement permettra également de favoriser une pratique agroécologique de l'élevage, respectueuse de l'environnement, du bien-être animal et garantissant une production de denrées de qualité.

Je suis saisi d'une demande de priorité de la commission sur l'amendement n° 408. Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

les objectifs et les moyens de notre politique de rénovation énergétique devaient être fixés par le Parlement dans une loi quinquennale. Nous aurions souhaité aller plus loin dans ce domaine, mais la nécessité d'obtenir un accord sur des sujets aussi sensibles et engageants nous a contraints à revoir certaines de nos ambitions. À l'occasion du vote de la loi de finances initiale, notre commission s'est alarmée de la réforme du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, qui s'est aux deux tiers de son montant et du nombre de ses bénéficiaires en un an. Nous avons adopté de premiers correctifs pour les ménages et pour les équipements éligibles, que le Gouvernement n'a pas retenus dans la version finale du texte.

de la loi Énergie-climat, nous attendons toujours la publication d'une dizaine de mesures réglementaires, d'une ordonnance et d'un rapport. Et pour ce qui est des crédits liés à la rénovation énergétique, il faut revenir sur la perte sèche de 400 millions d'euros induite par la dernière réforme du CITE ! Je crois nécessaire de desserrer très rapidement, mais temporairement, si vous le souhaitez, les conditions d'éligibilité à ce crédit d'impôt. Je me réjouis donc de cette proposition, initiée et défendue dans cet hémicycle dès le deuxième projet de loi de finances rectificative.

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les neuvième et dixième déciles, qui représentent les ménages les plus « aisés ». Une personne seule disposant d'un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n'a donc plus droit au CITE. De même, un couple avec deux enfants disposant d'un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n'a plus droit au CITE. On peut comprendre que le Gouvernement soutienne les ménages modestes et très modestes. Pour autant, en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les neuvième et dixième déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements. Le Gouvernement, qui pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an, a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone. Il est évident que les ménages modestes et très modestes, ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront, à eux seuls, relever ce défi.

près de 200 000 primes ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté. Il semble indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d'orienter les ménages, plus particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux neuvième et dixième déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d'efficacité énergétique des logements. La parole

Cet amendement de notre collègue Pascal Martin vise à rétablir une aide financière pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique plafonnée à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 euros par logement pour les équipements collectifs.

Le crédit d'impôt cinéma est un outil économique qui s'inscrit dans la politique du Gouvernement visant à relocaliser le tournage des films en France, tout en soutenant les industries techniques et l'emploi des techniciens en France. Il a été renforcé à plusieurs reprises dans le cadre des dernières lois de finances pour s'adapter aux besoins des producteurs d'oeuvres cinématographiques et gagner une vraie attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents.

pour les oeuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur les exercices 2020 et 2021.

Le crédit d'impôt international cinéma permet d'inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que leurs salaires et cachets sont fiscalisés en France grâce, notamment, à la retenue à la source. La limite globale de 30 millions d'euros par film reste inchangée. de proposer à ceux qui veulent tourner en France un marché gagnant-gagnant : l'élargissement de l'assiette par l'intégration des cachets étrangers, en contrepartie d'un paiement de l'impôt sur le revenu en France. Quel est l'avis de

Mme Catherine Dumas. Cet amendement vise à élargir le crédit d'impôt international cinéma aux films publicitaires. Les studios français sont soumis à une concurrence féroce de ceux, notamment, d'Europe de l'Est, qui cassent les prix. Avec les crédits d'impôt domestique en 2004, puis international en 2009, la France a commencé à relever la tête pour stopper la délocalisation et attirer les tournages étrangers, mais uniquement pour les films, à l'exclusion des films publicitaires. Ainsi, nombre de ces derniers échappent au tournage en France, profitant de rabais fiscaux à l'étranger. Étendre le crédit d'impôt international aux films publicitaires permettra à la France d'attirer sur son territoire des tournages synonymes d'emplois, de chiffre d'affaires et de recettes fiscales accrues.

Darcos. L'éditeur-distributeur est le maillon intermédiaire entre le producteur d'oeuvres cinématographiques et la salle de cinéma, entre le film et son public. Il assure l'édition, la promotion et la commercialisation des oeuvres. Il consent généralement une avance sur des films dont le succès en salle est très difficilement prévisible. Il n'a pas non plus la maîtrise de l'assiette de sa rémunération. Il s'agit donc d'un segment d'activité à risque. La fermeture des salles cinéma durant la crise sanitaire a mis à l'arrêt la principale activité et source de revenus des distributeurs, sans que les marchés secondaires viennent prendre le relais. Dans le contexte de réouverture des salles de cinéma, le risque financier pris par ces distributeurs est décuplé en raison des contraintes sanitaires- moins de séances, moins de sièges ... -et des incertitudes sur le retour des spectateurs en salles, dont la presse s'est fait l'écho aujourd'hui. Un crédit d'impôt en faveur des éditeurs de cinéma pour les dépenses d'édition et de communication dans des médias en France permettrait d'améliorer l'équation économique des distributeurs, sans distinction de genres cinématographiques et de taille d'entreprises. Ces dépenses pourraient bénéficier d'un taux dégressif au fur et à mesure de la reprise du marché

pour objet de permettre la prise en compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, au même titre que la stratégie nationale bas-carbone dans la stratégie de crise de l'État actionnaire, mise en oeuvre par l'Agence des participations de l'État, à travers le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État La PPE, qui constitue le document programmatique de référence dans le domaine de l'énergie, doit elle aussi être prise en compte : il s'agirait ainsi d'améliorer le contrôle du Parlement sur l'utilisation de ces 20 milliards d'euros d'aides, sans aller vers leur conditionnalité, peu adaptée aux réalités économiques. cela permettrait de crédibiliser, à un coût nul pour les finances publiques, les objectifs pris par l'État dans le cadre de la PPE, dont la réalisation est très attendue par les professionnels.

La transition écologique va demander énormément d'expertise et d'intelligence. Les services de l'État- le ministère de la transition écologique et ses opérateurs -devront jouer un rôle fondamental de bureau d'études et d'expertise pour les collectivités territoriales. Or, vous le savez, mes chers collègues, entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont fondu de 27 000 équivalents temps plein.

à entreprendre cette nécessaire conversion écologique si l'on diminue autant le nombre d'expertises dans l'administration centrale. Par ailleurs, nous sommes extrêmement inquiets de la diminution récurrente, drastique, pour ne pas dire infinie, des effectifs d'opérateurs essentiels comme Météo France,

Nous partageons l'avis du Gouvernement- c'est suffisamment rare pour être mentionné - : le CDD d'usage, c'est le contrat des surexploités. Or l'article 17 envoie un signal très clair : la crise justifie la précarisation maximale de l'emploi. La taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée dits d'usage était une incitation symbolique. Je ne suis pas certain que les entreprises aient renoncé à avoir recours à ces contrats en raison de cette taxe de 10 euros néanmoins le mérite de rappeler que les contrats courts doivent être plus chers pour les entreprises, afin de favoriser des recrutements en contrat de longue durée. Pour notre part, nous considérons que la précarité n'est pas une alternative au chômage ; seuls la formation et les emplois en CDI permettront de relancer le pays. Quel est l'avis de la commission

au patronat et aux organisations qui représentent les extras, qui sont dans une situation très difficile aujourd'hui- comme les intermittents, moins la compensation -, de continuer leurs négociations et de trouver une solution pour « déprécariser » ce travail.

les producteurs de gel hydroalcoolique, notamment, sont directement impactés par le présent article. On peut donc évidemment considérer qu'il a un lien avec la crise sanitaire actuelle et qu'il mérite d'être maintenu dans le présent projet de loi de finances rectificative. J'y insiste, il faut le maintenir.

un client qui revient ; un fraudeur qui trouve un système à frauder y revient également : c'est exactement ce qui se passe dans le cas du chômage partiel. Je vous propose donc, par cet amendement, que les demandes de versement d'indemnisation au titre du placement de salariés en position d'activité partielle s'accompagnent de la liste nominative des salariés visés, de leur identité, de leur numéro de sécurité sociale, ainsi que d'une copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cela me semble important.

incorrect, inapproprié pour des entreprises de bénéficier d'un soutien public à un moment où d'autres entreprises sont au bord de la faillite et ont vraiment besoin, elles, d'un accompagnement. La parole est à M. Jérôme Bascher,

Madame la ministre,

Il y a plusieurs formes de fraudes : celle qu'ont évoquée nos collègues Nathalie Goulet et Pascal Savoldelli sur les numéros Siret, par exemple, et une fraude massive sur le recours au chômage partiel pour les salariés. En l'espèce, je ne mets pas à égalité toutes les entreprises : je suis convaincu que certains petits chefs d'entreprise n'avaient jamais été confrontés à cette question et étaient persuadés qu'on pouvait recourir au chômage partiel et continuer à faire travailler ses salariés.

Vu l'ampleur de la fraude et des ramifications internationales révélées par les premières investigations, le parquet s'est saisi des dossiers au titre de sa compétence nationale en matière de lutte contre la criminalité organisée, d'autant que les virements étaient montés depuis l'étranger.

... Au cours des premières investigations, la justice a découvert des « demandes frauduleuses de versement d'indemnités » par télédéclaration, « en usurpant la raison sociale et le numéro d'identification Siret d'entreprises existantes qui ne demandaient pas à bénéficier

vise à raccourcir le délai dans lequel les Urssaf peuvent signaler aux cotisants la fin des contrôles non clôturés avant le 23 mars

un travers français -, on dégraderait encore la compétitivité de nos ports, sans que le produit de la taxe instaurée soit affecté à l'amélioration des infrastructures portuaires. Les préoccupations environnementales, notamment la qualité de l'air, peuvent être prises en compte par d'autres moyens, comme la modulation des droits de port pour les navires verts, le branchement des navires à quai ou la mise en place de zones de réduction des émissions des navires, comme celles que le Gouvernement promeut auprès de l'Organisation maritime internationale pour la Méditerranée. De telles mesures permettent de mieux répondre aux enjeux de nos ports.

préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en oeuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports., ce rapport est insuffisant, et la Cour des comptes l'a fait remarquer. Cet amendement vise à compléter ledit article, afin que le fameux rapport présente également les éléments synthétiques d'actualisation de l'étude d'impact du projet de loi devenu loi d'orientation des mobilités.

le texte un amendement équilibré répondant à la situation évoquée. Les copropriétaires seront indemnisés à hauteur de 70 % de la valeur vénale déterminée, abstraction faite du risque d'effondrement du bien concerné. Au-delà, sachez que nous nous attachons à préciser le cadre permettant de prévenir la survenue de telles situations ; des réponses pourraient notamment être apportées par le biais de projets de réaménagement globaux, qu'il s'agirait de mettre en place en amont. Dans ces circonstances, je vous propose de retirer cet amendement, au profit de l'amendement n° 1056

de 1 500 euros par foyer fiscal. L'objectif est d'allonger la durée de vie des produits, qui est un axe majeur de développement durable. Cela permettrait de favoriser, au moment de l'achat, les biens dont l'indice de réparabilité, créé par la loi Économie circulaire et qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2021, est élevé. Cet indice se transformera progressivement en indice de durabilité en 2024. Ce crédit d'impôt présenterait enfin l'intérêt de donner une bouffée d'oxygène au secteur de la réparation,

de l'environnement », d'un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés pour compenser 20 % des dépenses induites par la mise en oeuvre des préconisations de sécurité sanitaire. Cette mesure serait d'autant plus justifiée que le secteur du bâtiment, acteur incontournable de la transition énergétique, ne fait pas partie des secteurs bénéficiant de conditions d'accès privilégiées au fonds de solidarité à destination des entreprises,

naturel, applicable, notamment, au biométhane injecté dans les réseaux. Il s'agit de venir au secours de la filière française du biogaz, qui souffre des conséquences de la crise : 60 % des méthaniseurs étaient à l'arrêt fin avril, compte tenu de la baisse de consommation de gaz, mais surtout

d'un point essentiel, notamment au regard de la concurrence étrangère, qui ne concerne pas directement la crise, mais le plan de développement du réseau, qui doit se poursuivre. Ainsi, douze nouveaux établissements viennent d'être homologués au Liban, en Tunisie, aux États-Unis, au Laos, en Roumanie et en Ukraine. En comptant les extensions d'homologation, on atteint 5 000 élèves supplémentaires. L'Agence doit absolument pouvoir emprunter afin d'accompagner le développement de l'enseignement français à l'étranger,

les aides et secours

Les dossiers présentés pour l'obtention de ces bourses exceptionnelles sont très souvent rejetés sans que les raisons en soient données. Il paraît donc urgent de revoir les critères d'attribution en les adaptant au contexte local actuel et spécifique à chaque pays. Cet amendement a pour objet de permettre au Parlement d'exercer sa mission de contrôle de l'utilisation de l'argent public en demandant que soient rendus publics les critères d'attribution des bourses, que le Parlement soit informé des montants et des aides attribuées, ainsi que des refus et de leurs motifs. Lorsque la subvention destinée aux bourses n'est pas totalement consommée, c'est uniquement parce que les critères fixés par les administrations parisiennes ne tiennent pas compte des spécificités locales, différentes dans chaque pays. On peut donc se demander si la subvention exceptionnelle prétendument accordée n'est pas un leurre.

avec Jean-Yves Le Drian il y a une semaine, qui a accepté que son cabinet discute avec les élus des Français de l'étranger.

Le point de départ est l'indemnisation des propriétaires de la copropriété Le Signal. Cet amendement vise à donner une base législative pour sécuriser les modalités d'indemnisation des propriétaires de cette copropriété à hauteur de 70 % de la valeur vénale estimée, sans que soit pris en compte le risque d'effondrement.

les précédents amendements concernant Le Signal, cet amendement sera voté par l'ensemble de cette assemblée. Cela sera l'occasion de clore une histoire de six ans, faite de rebondissements et d'atermoiements. Des gens ont perdu du jour au lendemain leur lieu d'habitation et, depuis six ans, ils vont de procédure en procédure, avec toutes les angoisses et les inquiétudes que cela suscite. Il s'agit de familles modestes qui ont parfois dû être relogées

; l'attente était particulièrement forte. La perte de confiance qu'a mentionnée Mme Cartron s'est exprimée de façon douloureuse lors des rencontres que nous avons eues avec les riverains. Ce dossier doit en outre nous alerter sur la problématique de l'érosion de nos littoraux,

À ce titre, et au risque de sortir un peu du champ de l'article, j'aimerais appeler votre attention sur les besoins de la BITD, en particulier sur une entreprise française, Photonis, qui a aujourd'hui plus que jamais besoin de votre soutien. Il y a plusieurs semaines déjà, j'ai sollicité- en vain -un rendez-vous avec le ministre Bruno Le Maire pour évoquer ce dossier. Nous avons, en outre, échangé sur le sujet lors de votre audition devant la délégation sénatoriale aux entreprises. J'avais l'intention de faire passer deux messages clés. Contrairement à ce qu'indique le Gouvernement, il existe une solution alternative française à la vente pure et simple de Photonis au groupe américain Teledyne, mais aucun travail sérieux n'a été mené pour trouver et construire une telle alternative, le Gouvernement s'étant contenté de demander aux grands groupes du secteur s'ils étaient intéressés. Comme c'était prévisible, aucun d'entre eux ne l'est. De son côté le vendeur refuse d'ouvrir le dossier à d'autres parties potentiellement intéressées, tant que Teledyne est encore officiellement l'acheteur présumé. Or, je le répète, une solution alternative française existe, mais nécessite de regarder au-delà du simple cas de Photonis et d'avoir une vision stratégique et industrielle de la BITD. Faute de vouloir écouter un discours intelligent de stratégie industrielle, le Gouvernement s'apprêterait, si l'on en croit un article des de cette semaine, à autoriser la vente, en l'encadrant des précautions d'usage pour la protection des activités sensibles de l'entreprise et le soutien de l'emploi sur le territoire. L'objectif ne saurait être pourtant d'encadrer la vente de Photonis, mais bien d'arrêter et d'inverser un mouvement de fond qui fragilise la BITD en laissant partir progressivement les PME ou les ETI qui la constituent vers des actionnaires étrangers ou simplement opportunistes. Allons-nous abandonner à son sort une société emblématique du savoir-faire technologique et industriel français ? Allons-nous sacrifier l'intérêt général de la Nation au profit de l'intérêt particulier de quelques personnes privées ? Madame la ministre, nous sommes désormais dans l'urgence. Avant que l'irréversible ne se produise, je vous exhorte à trouver les moyens pour défendre la BITD et le temps de nous recevoir. La

qui ont pu survivre à la crise. L'urgence sanitaire a obligé certaines entreprises à réduire leurs effectifs, compliquant le respect des délais de greffage. Pour d'autres, les annulations de commandes les plongent dans le marasme économique et l'antichambre de la faillite. Pourtant, cette filière est est le leader mondial dans sa spécialité, avec 600 pépiniéristes et 230 millions de plants greffés,

n'ont pas pu faire appel au chômage partiel, donc à la solidarité nationale, n'ayant pas pu fermer.

pour les entreprises affectées par la crise sanitaire. Les services internationaux de transport de voyageurs ont été durement touchés par les restrictions de passages aux frontières. Ainsi, Eurostar n'a transporté que 0,7 % à 2 % des passagers transportés l'année dernière en avril et mai. Thalys, Thello et d'autres sont concernés. Malgré l'ouverture coordonnée des frontières intraeuropéennes depuis le 15 juin, le retour à la normale est beaucoup plus lent sur ces lignes que pour les services de transport régionaux ou nationaux ; il devrait prendre encore de nombreux mois. amendement vise à prendre en compte cette spécificité et à maintenir les conditions d'une concurrence équitable entre le transport aérien et le transport ferroviaire. Au regard des engagements environnementaux pris par la France et de la volonté du Gouvernement de favoriser une relance verte, rien ne justifie que le transport ferroviaire international ne bénéficie pas des mêmes dispositions que le transport aérien.

assez importantes et qui ne sont pas réservées au secteur aérien.

dès lors qu'elles ne bénéficient pas des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations salariales. Un certain nombre d'entreprises, qui ont pourtant été directement victimes des conséquences du covid,

pour l'exonération des charges sociales du 1 février au 30 octobre 2020 a été adopté en commission des finances. Le présent amendement a pour objet d'étendre cette modification aux collectivités de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes très impactées par la crise, dont les conséquences sur le secteur du tourisme vont continuer à se faire durement ressentir au moins jusqu'à la fin de l'année 2020.

s'agit d'un engagement financier extrêmement important offert par la collectivité aux entreprises. Nous avons eu d'autres débats sur des éléments de conditionnalité,

l'on peut admettre que, dans la précipitation, la panique et du fait du caractère totalement inédit de cette crise, certaines entreprises aient raté le coche de la publication de leur index au 1 avril,

que la crise ne remette pas en situation de citoyens de deuxième niveau les jeunes, les femmes, les seniors et un certain nombre de populations plus vulnérables, qui sont souvent les variables d'ajustement des crises. Monsieur Savoldelli,

économique. Les entreprises qui sont aujourd'hui les plus en difficulté vont devoir ajuster leurs sites. Une entreprise qui a perdu 50 % de son chiffre d'affaires

C'est la rémunération du salarié qui est versée. Certes, elle transite par l'entreprise, mais l'argent va directement au salarié et ne reste pas dans les caisses de l'entreprise au moment où celle-ci ne peut pas ou n'arrive pas à travailler.

n 33 rectifié et 34 rectifié ne sont pas soutenus. Madame la ministre, mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription le lundi 20 juillet, le matin, l'après-midi et, éventuellement, le soir de la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020. Acte est donné de cette demande. Nous siégerons donc demain, lundi, à moins que le rythme d'avancement de nos débats permette d'achever ce soir,